La séance est reprise, l'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finance adoptée par l'Assemblée nationale pour 2020 nous poursuivons l'examen au sein de la seconde partie du projet de loi de finances des différentes missions: le Sénat va examiner les crédits de la mission Justice une des sièges à terre des sièges. La parole est à monsieur Antoine Lefèvre, rapporteur spécial de la commission des finances, et vous avez 7 minutes chers collègues. Madame la présidente, mes chers collègues, Madame la Ministre, pardon, mes chers collègues, depuis plusieurs années, le ministère de la justice n'a pas les moyens d'exercer convenablement ses missions mais l'augmentation des moyens de la justice qui se matérialise depuis quelque temps, produit leur prendre ses effets dans les tribunaux, les établissements pénitentiaires les personnels expriment leurs difficultés, voire parfois leur désarroi pour exercer leur métier, ce qui n'est d'ailleurs pas sans conséquence sur leur état de santé, en effet, la surpopulation carcérale ou des délais de jugement trop long contribuent à décourager à décourager les agents qui parfois ne trouvent plus de sens à leur action, c'est dans ce contexte de fortes attentes et quelques mois après la promulgation de la loi de programmation 2018, 2 1000 22 et de réforme pour la justice que s'inscrit ce projet de loi de finances pour 2020, des attentes, s'agissant des moyens mais aussi en termes de fonctionnement de la justice, force est de constater que les crédits qui nous sont proposées aujourd'hui ne sont pas à la hauteur de ces attentes madame la Ministre, la commission des finances propose donc de ne pas adopter les crédits du ministère de la justice considérant qu'en dépit des transformations engagées, le gouvernement s'affranchit des engagements pris devant la représentation nationale, au moment du vote de la loi de programmation et de réforme pour la justice, avec un budget de 9,38 milliards d'euros en 2020, le ministère de la Justice bénéficieraient de 242 millions d'euros supplémentaires par rapport à 2019, soit une hausse de 2 7 pourcent de ses moyens, à périmètre constant. Mais alors que la loi de programmation votée par le Parlement en février dernier, prévoit une augmentation de 400 millions d'euros de crédits entre 2000 19 et 2020, le projet de loi de finances propose une hausse de près de 2 fois inférieur, or compte d'affectation spéciale Pensions les crédits augmentent de 2 8 pourcent soit 205 millions d'euros, cet écart résulte des crédits immobiliers de l'administration pénitentiaire ajusté au vu de l'avancement réel des opérations je m'interroge donc sur la sincérité de la programmation que nous avons adoptée puisque le gouvernement ne pouvait ignorer ces aléas, il y a 9 mois inhérents à la construction de prisons surtout cette révision à la baisse des crédits ne seraient pas rattrapé par la suite l'écart à la loi de programmation se porterait donc à 115 millions d'euros en 2022 40 pourcent de l'augmentation du budget de la mission est consacrée aux dépenses d'investissement dans la majeure partie concerne l'administration pénitentiaire, au lieu de construire 15000 places de prison sur le quinquennat 7000 places seront créées d'ici la fin du quinquennat et la construction de 8000 autres seraient lancés d'ici 2022, il est pourtant urgent de garantir un encellulement individuel et les conditions de détention digne, permettant également aux surveillants d'exercer convenablement leur travail s'agissant des recrutements, 300 des 1000 emplois créés en 2020, au sein de l'administration pénitentiaire permettrait de combler des vacances de postes de surveillants pénitentiaires jusqu'à présent, l'administration pénitentiaire, rencontrer des difficultés de recrutement, mais aussi de fidélisation des personnels, gageons que la réforme de l'organisation de la formation des surveillants pénitentiaires portera ses fruits, la prime de fidélisation prévus par le protocole d'accord signé en janvier 2018 a quant à elle, a été bien mise en oeuvre, mais il est encore un peu tôt pour en mesurer les effets, hors dépenses de personnel, l'augmentation des dépenses du ministère de la justice, de 3 pourcent s'explique actuellement par la nécessité de mettre à niveau l'informatique du ministère, le plan de transformation numérique poursuit sa mise en oeuvre ces investissements sont le signe du rôle crucial que le numérique doit jouer dans la modernisation de la justice. Il devra toutefois en résulter, à terme, la réalisation d'économies, il convient également de veiller à ce que la numérisation des procédures et des démarches demeure compatible avec un accès au droit sur l'ensemble des territoires afin que la fracture sociale et territoriale ne s'ajoute pas la fracture numérique, ce n'est pas le chemin que propose l'article 76 CS du PLF rattachés à la mission Justice qui prévoit une dématérialisation des demandes aide juridictionnelle, combinée à une suppression du bureau d'aide juridictionnelle dans certains tribunaux de grande instance, nous y reviendrons. Enfin, je terminerai en évoquant une inquiétude concernant le niveau des dépenses d'intervention de la mission dont la diminution résulte d'une baisse des moyens consacrés à l'aide juridictionnelle, en effet, la dépense relatives à l'aide juridictionnelle de 13 millions d'euros entre 2000 19 et 2020 grâce à une augmentation moins élevé de la dépense tendancielle et un transfert de 9 millions d'euros du Conseil national des barreaux, le gouvernement a toutefois profité de la budgétisation des ressources jusqu'ici affecté au Conseil national des barreaux d'un montant de 3 de 83 millions d'euros pour diminuer le montant des crédits budgétaires alloués à l'aide juridictionnelle. La dynamique de sa dépense qui résultent des réformes de 2015 et 2017 de mer en réalité identique dans le contexte de croissance dynamique de l'aide juridictionnelle, une révision de ses modalités de financement paraît indispensable mais la méthode proposée par l'article 76, terre des sièges du projet de loi de finances ne ne se veut pas être la bonne, nous en reparlerons tout à l'heure à l'occasion des amendements sur les articles rattachés à la mission Justice voilà, Madame la Ministre, les observations que je souhaitais faire sur ce projet de budget du ministère de la justice, que la commission des finances propose de rejeter, compte tenu du non-respect des engagements pris au moment du vote de la loi de programmation et de réforme pour la justice, je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le rapporteur, nous allons passer maintenant à monsieur Yves Detraigne, rapporteur pour avis de la commission des lois pour les programmes Justice judiciaire et accès au droit et à la justice pour 3 minutes. Merci madame la présidente, madame la garde des Sceaux, mais, mais, mes chers collègues, peu nombreux mais attentif, j'espère, les crédits de la mission Justice progresse de 2,8 pourcent en 2020, hors dépenses de pensions pour atteindre un montant total de 7,58 milliards d'euros de crédits de paiement, cela représente 205 millions d'euros supplémentaires mais l'évolution est moindre qu'en 2019 ou le budget avait augmenté de 4,5 parmi les programmes de la mission, le programme Justice judiciaire et celui qui augmente le mois l'effort consenti et seulement de 0,13 pourcent ce qui ne couvre même pas l'érosion liée à l'inflation, malgré tout, le renforcement des effectifs de magistrats se poursuit, le taux de vacance de poste n'est désormais plus que de 0 5 pourcent la situation est toutefois moins favorable pour les greffiers dont le même taux s'élève à 7 dans ce contexte, la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice implique la mise en oeuvre de nombreuses réformes d'organisation judiciaire, nous ne pouvons pas accepter que certaines se fasse selon des considérations électorales, malgré vos explications, madame la garde des Sceaux, la révélation par la presse d'une note de votre cabinet a jeté le trouble sur les conditions dans lesquelles la suppression de cabinet de juge d'instruction serait décidée par le gouvernement et sur l'objectivité des Chrysler retenus autre déception dans le budget, l'aide juridictionnelle,

s'il y ajoute une réforme adoptée dans la précipitation, à l'Assemblée nationale, alors que le gouvernement annonce un projet de loi sur ce sujet depuis plusieurs mois, si certaines des mesures proposées peuvent être intéressantes : elles sont pour moi invalidé par la méthode retenue qui est contestable, il s'agirait notamment de supprimer l'obligation d'avoir un bureau d'aide juridictionnelle dans chaque tribunal de grande instance, ce qui ne peut que susciter des craintes sur le maintien de l'accès à la justice pour nos concitoyens les plus vulnérables seraient également renvoyé au pouvoir réglementaire, la définition des plafonds d'admissions à l'aide juridictionnelle, or sans étude d'impact nul ne sait quel seuil envisage, envisage de retenir le gouvernement et quel sera le coût de ces mesures, je propose donc, comme notre collègue Antoine Lefèvre de supprimer cet article, compte tenu de ces observations. La commission des lois a donné un avis défavorable à l'adoption des crédits, des programmes de la mission Justice concernant la justice judiciaire et l'accès au droit, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à Madame Josiane Costes qui va s'exprimer en remplacement de Monsieur Alain Marc, rapporteur pour avis de la commission des lois pour le pour le programme Administration pénitentiaire et en sous son propre nom, en tant que rapporteur pour avis de la commission des lois pour le programme protection judiciaire de la jeunesse, dont vous avez. En tout, merci, madame.

dans une période où l'évolution des dépenses publiques et très contrainte, comme l'a expliqué la garde des Sceaux, cette hausse des crédits permettra de financer la création de milliers d'emplois et de poursuivre le programme de construction de nouvelles places de prison, avec l'objectif de livrer 7000 places d'ici la fin de l'année 2022, elle permettra aussi d'achever la montée en puissance du nouveau service national du renseignement pénitentiaire, créé en 2 1000 19 et de compléter les recrutements pour la nouvelle Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice toutefois la commission des lois, ne peut que regretter l'écart entre ce projet de budget la trajectoire fixée par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice, il manque environ 150 millions d'euros, alors que notre commission avait déjà jugé la programmation budgétaire insuffisantes au regard de l'ampleur des besoins, le gouvernement justifie cet ajustement à la baisse par le retard pris dans la mise en oeuvre du programme immobilier de l'administration pénitentiaire à l'approche des élections municipales, il deviendrait difficile d'obtenir l'accord des maires pour choisir le lieu d'implantation des futurs établissements il est vrai que nos concitoyens peuvent exprimer des réticences à l'idée que des personnes soient incarcérés près de leur lieu d'habitation, ce qui pose notamment un problème pour les structures d'accompagnement vers la sortie les sas que vous souhaitez à juste titre, implantés en centre-ville, près des services publics et des entreprises afin de faciliter la réinsertion des détenus, notre commission estime cependant que ces difficultés étaient parfaitement prévisible. Et qu'elles auraient donc pu être anticipé, elle considère également que ces 150 millions d'euros s'ils avaient été inscrits dans le budget aurait pu être utilisé pour financer des petits travaux de rénovation ou pour l'achat de matériel et d'équipements, ce qui aurait permis d'améliorer les conditions de travail du personnel ou de renforcer plus rapidement la sécurité des établissements pénitentiaires, qui reste pour nous un sujet de préoccupation constant, enfin, la commission des lois, s'interrogent sur la capacité du gouvernement à livrer les 7000 places dans le délai prévu, alors que l'agence pour l'immobilier de la Justice, rencontrent des difficultés pour recruter et fidéliser des professionnels qualifiés, c'est pour cet ensemble de raisons que la commission des lois a émis un avis défavorable à l'adoption des crédits de l'administration pénitentiaire pour 2020 nous ne sous-estimons pas le chemin parcouru depuis quelques années, mais il nous semble que l'incapacité du gouvernement à respecter dès la première année, la trajectoire budgétaire qu'il avait lui-même fixé, montre que l'effort réalisé n'est pas encore tout à fait à la hauteur des enjeux, je vous remercie pour votre attention programme protection judiciaire de la jeunesse, et là je me je m'exprime en mon nom propre, je reviens maintenant au crédit du programme protection judiciaire de la jeunesse, pour lesquelles la commission des lois a émis un avis favorable, celui-ci, la protection judiciaire de la jeunesse d'un budget de 736,6 millions d'euros hors pensions, soit une augmentation de 2,3 pourcent par rapport à 2019 il est marqué par la mobilisation pour préparer les réformes votées à venir, surtout la réforme de l'ordonnance de 1945 relative à la justice des mineurs dans l'entrée en vigueur est prévue au 1er octobre 2020, l'un des objectifs premiers de cette réforme et la réduction des délais de jugement des mineurs pour mettre en oeuvre cette mesure, le projet de budget prévoit la création de 70 équivalents temps plein, permettant de pourvoir 84 postes 94 postes d'éducateurs 24 postes étant créée suite à un redéploiement par ailleurs 5 emplois sont créés également par redéploiement pour favoriser la participation de la PJJ aux internautes complet, ce qui est très positif, or personnel le budget de la PJJ continue sa progression entamée il y a 3 ans, avec une augmentation de 3 pourcent cette augmentation se répartit entre le secteur associatif habilité SH dont le rôle est croissant et le secteur public, si l'on ne peut que se féliciter de ces augmentations qui paraissent nécessaires au moment où la PJJ recrute et ce, avec difficulté, de plus en plus d'éducateurs contractuels, on peut s'interroger sur les ondes, pas les orientations retenues à moyen terme en effet la création des postes d'éducateurs dans le projet de budget correspond à : renforcement du secteur ouvert mais le contexte général est celui d'un d'un d'un recours accru au secteur fermé, c'est-à-dire privative de liberté pour les mineurs, il me paraît important d'insister sur le fait que l'importance accordée au centre éducatif éducatif fermé comme structure et au secteur associatif habilité comme opérateur ne doit pas aboutir à détourner la PJJ de sa vocation première, l'éducation et l'insertion des jeunes en danger en s'appuyant sur les compétences des équipes éducateur spécialisé et en milieu ouvert, j'en viens maintenant au sujet que la commission des lois, cette année, l'incarcération des mineurs en juin dernier un pic de 894 mineurs incarcérés a été atteint, renouant avec les chiffres de la fin des années 80 au total plus de 3000 mineurs sont incarcérés, chaque année, une catégorie de jeunes, en particulier les mineurs non accompagnés est surreprésenté en prison, ils occupent un tiers des places pour mineurs de Fleury-Mérogis il fraude, il faudra donc madame la ministre nous pencher sur le traitement pénal dont ils font l'objet, mes déplacements m'ont conduite à étudier plus pas plus particulièrement la situation de l'Île-de-France, cette région qui est celle qui compte le plus grand nombre de mineurs incarcérés nécessite la création d'un nouvel établissement carcéral pour les mineurs, vous nous avez indiqué madame la garde des Sceaux, que l'établissement de mots connaît qui avait été établi initialement prévu, conçu comme un établissement pour mineurs sera simplement doté d'un nouveau quartier pour mineurs, ce qui signifie que le taux d'encadrement sera moindre, c'est un choix décevant au regard des besoins des mineurs en termes d'accompagnement, d'éducation et d'aide à l'insertion, on ne peut par contre que ce fait, les que le quartier pour mineurs de Fleury-Mérogis de Fleury-Mérogis bénéficiera bien d'un bâtiment dédié, même si tout reste à construire pour conclure sur ce point précis des mineurs détenus les efforts en terme d'éducation doivent être accentuée ce qui relève de l'Éducation nationale et la PJJ doit trouver pleinement sa place en milieu carcéral, notamment dans les établissements pour mineurs afin d'assurer la continuité de la prise en charge des jeunes pour lesquels l'incarcération reste une mesure exceptionnelle. Je vous remercie. Merci dans la suite de notre discussion, je vous rappelle que le temps de parole attribués à chaque groupe pour chaque unité de discussion qu'on prend le temps d'intervention général et celui de l'explication de vote par ailleurs le gouvernement dispose au total de 20 minutes pour intervenir et la parole est à monsieur Emmanuel Capus pour le groupe, les indépendants, qui est prêt pour 6 minutes de temps de parole. Merci madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des finances, Madame et messieurs les rapporteurs spéciaux et pour avis, mes chers collègues, le projet de loi de finances pour 2020 prévoit une augmentation des crédits et des employes de l'ensemble des programmes de la mission Justice ce qui en soi est une bonne nouvelle, le montant des crédits demandés pour 2020 atteint ainsi près de 9 milliards d'euros en autorisations d'engagement et 9,4 milliards d'euros en crédits de paiement, le plafond prévisionnelle de l'emploi déplace légèrement les 88000 équivalents temps plein travaillés, ce qui correspond à un relèvement de 1520 employes de l'autorisation de recrutement. Si cette évolution des crédits et des emplois est positive, elle marque en revanche un décrochage par rapport aux engagements pris dans le cas de la loi de mars 2019 de programmation pour 2018, 2 1000 22 et de réforme pour la justice, celle-ci prévoyait pour l'exercice 2020 la création de plus de 1620 emplois et l'inscription en loi de finances initiale de près de 400 millions d'euros supplémentaires en crédits de paiement. Cette progression des crédits et des emplois apparaît modeste au regard des efforts nécessaires au redressement de la justice, ce qui se trouve toujours, qui se trouve toujours pardon dans une situation critique, tant au niveau de ces délais que de ses moyens. Ce constat : notre groupe parlementaire l'avait déjà dressé en 2018 et en 2019 à cette même tribune. Je souhaite, Madame la Ministre, plus particulièrement, formuler des observations spécifiques à 2 des 3 programmes de la mission Justice tout d'abord s'agissant des moyens dévolus aux juridictions judiciaires, notre groupe, notre groupe, comme l'an dernier, regrette que ce budget soit celui qui augmente le moins parmi tous les programmes de la mission Justice en effet l'effort consenti est de seulement 0,13 pourcent ce qui ne permet pas de couvrir l'érosion liée à l'inflation. Néanmoins, il faut saluer la poursuite du renforcement des effectifs des juridictions, avec la création nette de 384 emplois en 2020 et la quasi-résorption du taux de vacance de postes de magistrats, tout comme celle de l'augmentation des crédits en faveur du numérique, de l'ordre de 7 Mais toutes ces mesures ne doivent pas occulter une situation qui demeurent malheureusement préoccupante dans les juridictions, avec des délais de traitement qui s'allonge et une situation chronique de sous-effectifs lié aux vacances de postes de greffiers. Il en va de même de la progression des crédits du programme consacré à l'administration pénitentiaire, en effet, cette progression est réel et appréciable, même si elle demeure inférieure d'environ 150 millions d'euros à celles prévues par la loi de programmation. Un autre point positif doit être relevé, il s'agit de l'augmentation des effectifs, avec la création de 1000 postes je crains néanmoins que, compte tenu du nombre élevé de personnes placées sous main de justice et des sous-effectifs chroniques constatés ces créations d'emplois ne suffisent pas à améliorer les conditions de travail des personnels, en effet, l'administration pénitentiaire, comme de nombreux autres administrations rencontrent des difficultés de recrutement, avec sans doute une difficulté supplémentaire lié aux conditions de travail très rude propres à ce milieu. Enfin, le programme immobilier doit matérialiser l'engagement présidentiel de construire 15000 places de prison avant la fin du quinquennat Je crois avoir bien compris ce ce ce chapitre il sera séquencé en 2 livraisons successives 7000 places doivent être livrés avant la fin de 2000 et le 8 1000 autres entamé avant 2022 pour une livraison effective avant la fin de l'année 2027, vous savez, madame la ministre, que je me réjouis à cet égard, de l'engagement que vous avez pris d'y faire figurer un nouvel établissement pénitentiaire à Trélazé dans le vous savez et vous connaissez bien la maison d'arrêt d'Angers et vous connaissez son état totalement déplorable. Mes chers collègues, nous le savons tous la situation que vivent les personnels dans les établissements pénitentiaires et dramatique, notamment face à la hausse du nombre de personnes placées sous main de justice notre groupe serait donc très favorable à une augmentation des crédits au regard des enjeux auxquels notre justice doit faire face aussi, pour l'heure, le groupe les indépendants demeurent vigilants concernant les crédits de la mission Justice du projet de loi de finances pour 2020, je vous remercie. Merci, la parole est maintenant à monsieur Jean-Pierre Sueur pour le groupe socialiste et républicain et vous avez 10 minutes.

madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues. Le coup de la justice, si l'on peut dire par Français. C'est 65,90 euros par an. Pour les Allemands, les Britanniques, ces 122 euros. Par habitant et par an. D'après une étude que vous connaissez bien du Conseil de l'Europe, la France est au 37ème rang sur 41 sachant de son budget de la justice, s'agissant notre pays contre compte 4 fois moins de procureurs que la moyenne européenne 2 2 fois moins de juges et 2 fois moins de personnel de greffe par habitant. Certes, face à ces faits, il est clair que le budget de la justice est en constante augmentation depuis 2002. Soit, depuis plus de 15 ans. Et pourtant, l'écart reste toujours très important. Et pourquoi, hé bien parce que les augmentations décidées, année après année, porte sur un budget historiquement tellement bas que le regard que le retard structurel n'est jamais rattrapé. Alors Madame la Ministre, c'est à l'aune de ces constats, qu'il faut parler de votre budget est certes. J'ai bien dit. Que l'effet que j'ai rappelées concerner tous les gouvernements depuis longtemps. Ce qui nous manque et combien de fois et Jules, occasion de le dire à cette tribune, mes chers collègues, et avant, à l'Assemblée nationale. Il y a longtemps. C'est une véritable loi de programmation. Qui s'imposerait en quelque sorte à tous les gouvernements. Nonobstant les principes de l'annualité budgétaire. Et qui ferait. Que. L'on ferait un effort très considérable pour enfin rattraper le retard. Vous nous direz qu'il y a une loi de programmation qui a été inscrite dans la loi de réforme de la justice que vous nous savez. Celle-ci prévoyait la création d'emplois et il y a des emplois. Ils sont créés c'est vrai. Toutefois, nous sommes navrés de constater. Que malheureusement les crédits qui été promis. Qui était programmé dans cette programmation ne sont pas présents au rendez-vous. Ainsi, il manque au bas mot. 150 millions de crédits cette année. Par rapport à ce que vous-même aviez proposé d'inscrire dans la loi, cette loi de programmation ou cette loi de réforme de la justice est ce que le le le Parlement avait accepté. Et non seulement acceptée mais souhaitée, nous avions d'ailleurs souhaité davantage. Plusieurs constatations aujourd'hui. Apparaissent une baisse de 45,6 pourcent des investissements pour la justice judiciaire. Une baisse de 3,35 pourcent du fonctionnement de l'administration pénitentiaire, une baisse de 2,5 pourcent de la conduite, et du pilotage de la politique de la justice, une baisse de 20 pourcent pour l'accès le support à l'accès au droit et à la justice, d'autre part pour ce qui est des places de prison. Je tiens à souligner. Que celle-ci, bien entendu, bénéficient de crédits en augmentation, comme d'ailleurs l'ensemble de l'administration pénitentiaire. Des postes vont être créés, mais souvent, ces créations de postes vont permettent de combler les vacances qui sont également très nombreuses, mais vous le savez madame la Ministre, il n'y a jamais eu autant de personnes incarcérées en France et la France est le seul pays européen où le nombre de détenus augmente dans ces proportions, ce nombre, il a atteint un nouveau record avec 71828 personnes détenues au premier avril 2019, ce qui pose à nouveau avec une acuité toute particulière, la question de la mise en oeuvre efficace et effective des alternatives à la détention, sujet sur lequel les nécessaires réponse ne nous paraissent pas être au rendez-vous quand on voit cette surpopulation qui appellerait l'augmentation sensible de ces mesures. J'ajoute que, pour ce qui est des mesures annoncées lors du Grenelle des violences conjugales auxquelles vous savez participé Madame la Ministre, nous pouvons craindre que les crédits qui sont annoncés ou qui sont supposés sont inférieurs aux besoins qui apparaissent pour lutter efficacement contre les violences faites aux femmes. J'ajoute que, pour ce qui est de la l'accès à la justice et de l'aide juridictionnelle, il y a une remise en cause avec une baisse des crédits qui diminue de près de 22 millions d'euros en 2020. Alors je sais que l'Assemblée nationale a voté des dispositions par rapport à l'aide juridictionnelle, mais nous sommes très sceptiques et même plus que sceptique par rapport à ces dispositions. Premièrement, il ne nous paraît pas justifié. De prendre le revenu fiscal de référence. Comme indicateur alors qu'aujourd'hui, tous les revenus de toutes natures sont prises en compte. Nous ne sommes pas favorables à la suppression de l'obligation dans chaque TGI d'un. D'un bureau de l'aide juridictionnelle, d'un point d'accès à l'aide juridictionnelle. Et d'autre part, nous ne pensons pas qu'il soit justifié d'écarter un certain nombre de public en vertu de ce qui est appelé une politique uniforme du bureau d'aide. Juridictionnel, nous pensons qu'il faut rester très s'attentif aux besoins d'aide juridictionnelle et naturellement, ce budget ne répond pas à cette question puisqu'il diminue les crédits pour l'aide juridictionnelle. Je voulais aborder, a encore d'autres 2 autres points le 1er, celui de la spécialisation, madame la ministre, vous avez dit ici même au Sénat. Que pour la spécialisation des tribunaux dont certains craignent qu'elle soit en fait une disposition. Qui d'une certaine manière pallierait à l'idée de supprimer été juridiction on maintiendrait, vous avez dit hautement qu'on maintiendrait toutes les juridictions mais si certaines. Sont déchargés d'un certain nombre de prérogatives, naturellement, cela peut poser des problèmes, et vous avez dit que rien ne saurait être imposé. Que tous ceux qui seraient faits serait appelée par les juridictions elle-même, or quand on se trouve dans une circonstance madame le Garde des Sceaux, je connais un département c'est celui où je suis élu, où il y a 2 tribunaux de grande instance ou lorsque l'on consulte les représentants des magistrats. Des personnels des avocats. Il n'y a pas d'accord sur. Certaine mutualisation spécialisations qui sont proposées est ce que vous pouvez confirmer que, dans ce cas, hé bien on restera dans l'état actuel des choses, puisque vous en avez pris l'engagement ou est-ce que vous pensez que cela pourrait être remis en cause si, par exemple, des chefs de cour, aller à l'encontre, je ne l'imagine pas de ce que pensent l'ensemble des magistrats, l'ensemble des personnels ou des avocats. Et puis comment ne pas revenir Madame le Garde des Sceaux sur cette affaire qui nous a beaucoup émues ici au Sénat. Le fait que soit publiée une note de votre ministère qu'elle soit parue dans la presse indexant en quelque sorte l'éventualité de décision quant à l'affectation des juges d'instruction à leur maintien ou à leur suppression sur telle ou telle considération électorale, vous savez que je vous ai beaucoup interrogé là-dessus que je vous ai posé des questions très précises auxquelles vous avez toujours répondu par un mutisme tenace, je dois le dire, et cela crée un contexte qui n'est pas non plus favorable alors pour toutes ces raisons. En dépit des efforts qui sont faits. Et que je tiens ça souligné puisque les crédits sont en augmentation, en dépit des efforts qui sont faits pour toutes les raisons que je viens d'énumérer notre groupe ne pourra pas voter les crédits que vous nous présentez pour cette année 2020, je vous remercie. Merci, la parole est maintenant à monsieur Thani Mohamed Soilihi pour le groupe La République en marche. Pour 7 minutes. Madame la présidente, madame la garde des Sceaux, monsieur le rapporteur général madame et monsieur les rapporteurs pour avis, mes chers collègues, pour la 3ème année consécutive, le budget pour la justice connaît une nouvelle augmentation de ces crédits, en effet, après une hausse significative de 3,9 pourcent en 2018 le budget s'élève pour l'année 2020 à 7,6 milliards d'euros, ce qui représente une progression de près de 4 pourcent soit 300 millions d'euros supplémentaires, on peut choisir de voir le verre à moitié vide et de dire que, malgré une hausse des crédits consacrés à la justice, ces derniers restent proportionnellement bas par rapport à d'autres missions et n'atteignent pas le niveau de ceux accordés par nos voisins européens, c'est ce que notre collègue sur vient de dire, on peut dire aussi que cette hausse est inférieure à la trajectoire qui était fixé dans la loi de programmation budgétaire 2018, 2022 adopté en février dernier, qui aurait dû être de 5 mais comme vous nous l'avez expliqué madame la garde des Sceaux, le budget a été revu à la baisse en raison de retards, l'un des chantiers de projet immobilier pénitentiaire et ça c'est quelque chose de factuel, à l'inverse, nous avons décidé de voir le verre à moitié plein et de constater sans satisfecit excessif car il y a beaucoup encore beaucoup de chemin à parcourir pour mettre la justice un niveau dans notre pays, nous pouvons constater tout de même que l'évolution depuis 2013, des moyens globaux alloués à la justice judiciaire montrent une hausse significative, on peut également se réjouir de l'augmentation réelle des effectifs présents un juridiction avec ce budget, ce sont 1520 emplois qui seront créés, ce qui portera, vous l'avez rappelé madame la garde des Sceaux à 3920 le nombre d'emplois créés depuis 2018, l'administration pénitentiaire bénéficiera donc d'un millier de postes supplémentaires et de près de 84 millions d'euros dédiée aux programmes immobiliers qui permettront de tenir compte des revendications légitimes des surveillants pénitentiaires et d'améliorer le fonctionnement et la sécurité des établissements dans lesquels ils travaillent, les effectifs de magistrats sont également renforcés dans les juridictions, avec la création de 384 emplois afin de poursuivre le véritable effort de réception du taux de vacance de postes de magistrats entrepris par le gouvernement, la protection judiciaire de la jeunesse profitera aussi de cette augmentation en moyens humains et se verra doté de 94 postes d'éducateurs, de plus, le ciblage de 70 emplois de magistrats et de 100 emplois de greffiers, la poursuite de la diversification de la prise en charge des mineurs délinquants, la construction de centres éducatifs fermés et la rénovation du parc immobilier permis grâce au crédit du 17 millions d'euros concourront à la prochaine mise en oeuvre de la réforme de la justice pénale des mineurs, qu'il a un truc en vigueur au 1er octobre 2020. Ces créations d'emplois permettront également aux juridictions et au service pénitentiaire d'oeuvrer dans le sens de la diversification des peines et du développement des alternatives aux peines de prison qui faisait l'objet de l'un des 5 objectifs prioritaires de la loi de programmation 2018, 2 1000 22 et de réforme de la justice, du 23 mars 2019, je pense notamment au bracelet antirapprochement qui permettrait de géolocaliser et maintenir à distance les conjoints et ex-conjoints violents et dont le périmètre d'éloignement serait fixée par un juge, il me semble tout aussi important de souligner que ce budget consacrent des moyens conséquents pour poursuivre la modernisation numérique de la justice, vous nous avez assuré Madame la Garde des Sceaux, que les réseaux haut débit serait effectif sur un millier de sites judiciaire fin 2020, y compris en Outre-mer, j'y veillerai, car dans ces territoires où l'insularité et l'éloignement géographique complexifie grandement l'accès au droit, cette transformation numérique et capital, je dirais, un dernier mot sur l'aide juridictionnelle, qui à mon sens, nécessiterait une réforme d'ampleur et qui pourtant vient de faire l'objet de modifications aux conséquences importantes mais incertaine faute d'étude d'impact, à l'Assemblée nationale, ces modifications suscite évidemment des interrogations, quel sera l'impact du nouveau critère de revenu fiscal de référence par rapport à l'ancien critère de ressources de toute nature sur le périmètre des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, les dispositions nouvelles ne sont-ils pas, ne sont-elles pas entaché d'incompétence négative et dans ce cas-là, n'y a-t-il pas un risque d'inconstitutionnalité, autre interrogation : l'implantation des bureaux d'aide juridictionnelle au sein des tribunaux de grande instance date de 1851 le renvoie à un décret pour les futures implantations inquiète la profession d'avocat, sans garantie du principe de l'existence d'un but d'un barrage dans le ressort de chaque cour d'appel ne serait-il pas, par ailleurs préférable de prévoir que le décret soit pris en Conseil d'État, en conclusion, nous pensons qu'avec cette progression des crédits, le gouvernement confirme la priorité accordée à la justice de notre pays, ce budget consacrent un effort particulier aux dépenses de personnel et d'Aventis d'investissement dans notre justice a cruellement besoin, c'est la raison pour laquelle, nonobstant les interrogations dont j'ai fait écho et j'espère Madame la garde des Sceaux, que vous nous apporterez des réponses, c'est la raison pour laquelle, malgré tout, le groupe La République en marche votera en faveur de ces crédits. Merci, la parole est maintenant à Madame Éliane Assassi pour le groupe CRCE pour 6 minutes de temps de parole. parole. La présidente, madame la garde des sceaux, Madame et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je dirais que cette mission a quand même ceci de, de, de, de particulier, c'est que la mise en oeuvre et de la loi de programmation 2018, et de réforme pour la justice, récemment adopté ont déjà fixé le plafond de dépenses qui se qui seront consacrés chaque année à la mission Justice ainsi, il est prévu d'atteindre à l'horizon 2022, un budget de 8,125 milliards d'euros hors contribution au compte d'affectation spéciale Pensions, peu de surprises, donc à la découverte de ce budget en augmentation comme prévu et qui suit peu ou prou les orientations annoncées que nous contestions déjà lors de la discussion de la dite réforme seulement alors que la loi de programmation pour la justice, prévoyait une augmentation de 400 millions d'euros, Madame la Ministre, vous ne vous ne proposez finalement que de lui affecter 200 millions l'an prochain, pourtant je voudrais rappeler, comme l'a fait Jean-Pierre Sueur, que le système judiciaire français est l'un des plus mal dotées en France, le rapport 2018 de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice décrivait d'ailleurs le système judiciaire français comme l'un des plus mal dotées parmi les États du Conseil de l'Europe, tant en terme de budget consacré à la justice que d'effectifs, de magistrats, avec 13 magistrats et 47 personnels judiciaires pour 100000 habitants contre 31 et c'est son 5 pardon pour la médiane européenne ainsi alors que pour 2020 le nombre d'emplois créés, présentée comme un effort considérable avec un rythme de 100 postes de magistrats en plus par an, il faudrait plus d'un siècle à la France pour rejoindre la médiane des États du Conseil de l'Europe, s'agissant des tribunaux de grande instance leur activité ne réduise ne ne réduisant pas et les créations de postes étant insuffisantes leur délai moyen de traitement n'ont fait qu'augmenter depuis maintenant plusieurs années, dans ce cadre, je ne peux Madame la Ministre que réitérer notre inquiétude quant à la mise en oeuvre et de la loi de programmation 2018, 2 1000 22 et de réforme pour la justice, qui entraînera notamment la fusion du tribunal d'instance et de grande instance au sein du tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, comme le relève le syndicat de la magistrature, la disparition de cette juridiction, et par conséquent de ses moyens propres ne pourra qu'avoir un n'est pas un impact négatif sur le délai moyen de traitement des affaires qui relevait de sa compétence, dès lors que ces moyens seront mutualisés avec l'actuel TGI dont les délais sont catastrophiques en outre la disparition des tribunaux d'instance, marquera un recul frappant pour notre pays en matière d'accès aux juges reculent alimenter d'ailleurs par le déploiement de la visio-conférence des moyens en plus pour cette mission, certes, mais au profit d'une justice déshumanisée, très peu pour nous avec l'augmentation de 20 pourcent du parc de visioconférence, le principe de la présence physique du justiciable à l'audience, semble donc devenir marginal par rapport à celui de l'audience par visioconférence, nous dénonçons régulièrement cette évolution majeure de la procédure pénale, la visioconférence ne permet ne permettant ne permettant pas un exercice réel des droits de la défense pour le justiciable et compliquant le déroulement de l'audience, outre le recul en matière d'accès aux juges, porté par la volonté des temps de la visioconférence, un autre principe, celui de l'incarcération à Touba illustrent ce budget malgré un affichage politique contraire ainsi 159 emplois sont réservés aux ouvertures d'établissements pénitentiaires et 83,5 millions d'euros sont consacrés aux crédits immobiliers, soit une augmentation de 27 pourcent par rapport à 2019, l'objectif affiché est ainsi la création de 15000 places de prison supplémentaires à l'horizon 2025, alors bon, si des collègues sénatrices et sénateurs regrette au-delà même de la majorité sénatoriale, le manque d'ambition en la matière, nous nous inquiétons pour notre part du tout à l'inverse que ce budget soit presque totalement dédié à l'enfermement d'autant plus que cette logique délétère de priorisation de l'enfermement est aussi coûteuse qu'inefficace en termes de prévention de la délinquance, la même logique et pourtant également retenu en matière de protection judiciaire de la jeunesse, l'augmentation des crédits et des effectifs de ce programme étant presque entièrement absorbé par la construction de 20 nouveaux centres éducatifs fermés, or, là encore, nous maintenons notre opposition à la création de ces nouveaux centres éducatifs fermés qui n'ont d'éducatif que leur nom à l'inverse, nous prenons une revalorisation urgente du budget concernant le suivi des mineurs en milieu ouvert, enfin concernant l'aide juridictionnelle, là encore, les apparences sont trompeuses, puisque le projet de loi de finances, laisse apparaître une augmentation des crédits qui seraient consacrés à l'aide juridictionnelle, alors qu'en réalité il n'en est rien, en effet, comme le dénonce, là aussi, le syndicat de la magistrature, je cite cette augmentation est uniquement due à l'intégration dans les recettes de crédit qui était auparavant affecté au Conseil national des barreaux, il s'agit donc uniquement d'un changement de périmètre à périmètre constant, c'est en réalité une baisse de 3,2 pourcent du budget consacré à l'aide juridictionnelle, qu'il faut constater, se situe largement en dessous de la moyenne européenne pour le budget par habitant alloués à l'aide juridique, on assiste donc à une diminution de ce budget, qui sacrifie une politique publique pourtant crucial pour l'accès de tous à la justice, y compris les plus démunis et des conditions de rémunération décente des avocats, qu'il est défendu, donc vous aurez compris pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce budget qu'il serait urgent d'abonder, madame la ministre, à la hauteur de l'enjeu de missions de service public que représente notre justice, dans l'intérêt de tous les justiciables, mais aussi dans l'intérêt de notre état de droit, je vous remercie. Merci, la parole est maintenant à Madame Sylvie mais vermeil et pour 8 minutes.

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, Madame et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le budget 2020 de la justice présente des évolutions positives, il peut ainsi paraître surprenant que pour la première fois au cours des dernières années, aussi bien notre commission des finances que notre commission des Lois propose de ne pas adopter les crédits de la mission Justice c'est une première et cela est-il justifié, je souhaite donner premièrement notre analyse du budget 2020, deuxièmement exprimé certains doutes troisièmement conclure par nos points d'attention le budget 2020 comporte des évolutions positives que nous saluons, même si le Graal de la trajectoire fixée par la programmation pour la période 2018, 2022, que nous avons adoptée récemment, n'est pas atteint. On remarque que le budget est en augmentation de 4 pourcent que plus de 1000 500 emplois vont être créés qu'une inscription de l'intégralité du financement de l'aide juridictionnelle, redonnant au budget, une sincérité de bon aloi que la vacance des postes de magistrats problème, problème récurrent et ramenée à un taux de 0 9 pourcent ce qui est une très bonne nouvelle ce résultat satisfaisant n'avait certainement pas été atteint depuis très longtemps 161 millions de crédits de paiement sur la programmation immobilière judiciaire et enfin, plus 400 emplois au service des services au bénéfice des services d'insertion et de probation, les CPIP, l'application des peines, talon d'Achille de la justice n'est plus le parent pauvre et nous a, que nous avons connu longtemps on peut relever la création des 145 emplois en vue de l'ouverture à venir de places de prison ainsi que la forte augmentation des crédits en faveur de la sécurité pénitentiaire deuxièmement nos doutes que je citerai dans le désordre : tout d'abord la création du Parquet national antiterroriste que vous mettez en avant. Nous ne sommes pas convaincus d'une amélioration par rapport à la compétence antérieur du parquet de Paris et l'efficacité que celui-ci pouvait trouver dans une mobilisation rapide de magistrats en nombre, la création de l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice, notre groupe a peu d'appétence pour la multiplication des agences les EPM les établissements pour mineurs nous semble connaître beaucoup de dysfonctionnements, nous ne demandons pas à leur suppression mais a minima votre vigilance particulière, troisièmement, je vous présente nos points d'attention en conclusion l'année 2020 sera-t-elle l'année de la réalisation et des premiers résultats, comme vous vous plaisez à le dire. Nous le souhaitons, mais ne croyons pas que tout soit une question de budget où passe par une réforme de la justice, nous ne pensons pas que la justice doivent se complaire dans les grands principes, les grands débats de société où les assauts intellectuel qui rivalisent de brio, à l'occasion des discours de rentrée, notre groupe pense que la justice a besoin d'humilité et de ténacité, d'un effort du quotidien, pour paraphraser l'image chère à nos collègues de la commission de la Défense à propos d'une loi de programmation militaire à hauteur d'homme, nous souhaitons une justice à hauteur d'homme sans vouloir réduire le prestige attaché à votre mission Madame le Garde des Sceaux, nous sommes convaincus que votre ministère a besoin d'une culture du management, une culture de la gestion des ressources humaines, une culture du pilotage transversale des projets qu'ils soient immobilier ou informatique pour symboliser notre approche, nous pensons plus utiles au fonctionnement de la justice d'avoir une chaîne pénale informatique fluide de la plainte au jugement et à son exécution fluide pour les policiers, les greffiers, les magistrats, les avocats tous les auxiliaires de justice ou encore les victimes que de débattre indéfiniment de réforme pénale, la justice est pour nous très représentative du fonctionnement en silo de notre pays. Le budget que vous nous présentez permet des avancées, si elles étaient accompagnées d'une plus grande horizontalité de votre ministère, notre groupe y verrait une oeuvre très utile en conclusion et pour répondre à la question que je posais au début de mon intervention, les critiques multiple qu'ont détaillé nos collègues rapporteurs sont telles que nous ne pouvons soutenir ce budget Madame la garde des Sceaux, j'ai rappelé un certain nombre d'avancées, mais le fait qu'un budget augmente ne suffit pas à démontrer que l'effort soit à la hauteur des enjeux, je terminerai en reprenant un point cité par mon collègue Yves Détraigne oui, le budget des juridictions judiciaires augmente mais l'effort consenti ne permet même pas de couvrir l'érosion liée à l'inflation, suivant l'avis de notre commission des finances et de notre commission des lois, le groupe Union centriste votera contre les crédits de la mission Justice je vous Rehmer.

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, l'examen de cette mission justice doit nous amener à nous pencher, à la lumière des problématiques auxquelles la France face aujourd'hui sur la question centrale de la protection judiciaire de la jeunesse et mes propos concerneront particulièrement la PJJ alors que des phénomènes de délinquance, ils viennent en plus en plus précoce chez certains jeunes, notre pays doit assurer une protection judiciaire de la jeunesse, efficace et dotée de moyens et de d'ambition pour 2020, le gouvernement propose d'augmenter de 2 pourcent les crédits du programme 182 protection judiciaire de la jeunesse, soit 18 millions d'euros, dont 8 millions de masse salariale, ce projet de loi de finances pour 2020 prévoit donc, comme cela a été dit, la création de 70 équivalents temps plein d'éducateurs supplémentaires, selon la protection judiciaire de la jeunesse, ces nouveaux postes seront essentiellement consacrés à la prise en charge éducative en milieu ouvert, dont les effectifs actuels sont gravement insuffisants, notamment pour permettre une prise en charge socio-éducatives efficaces afin de repérer au plus vite les mineurs en risque de réitération de décrochage scolaire ou de rupture familiale et de travailler avec leur famille néanmoins un problème de taille demeure intactes, celui de la qualification et de l'expérience des éducateurs, malgré les efforts affichés en terme de recrutement d'éducateurs, il ne suffit effectivement pas de créer des postes supplémentaires, en effet, comme tout comme la problématique existent au niveau de l'Éducation nationale pour les enseignants débutants nommés dans les quartiers les plus difficiles, il est nécessaire est crucial de mener une réflexion sur l'expérience des éducateurs qui doivent être suffisamment armés pour encadrer les jeunes qui leur sont confiées, une formation solide et complète permet d'éviter d'entraîner un turn-over excessif dans les équipes et de mettre en difficulté ces éducateurs au tout début de leur carrière, que ce soit en milieu ouvert ou dans les centres éducatifs quant aux centres éducatifs fermés, un programme de création de 20 des établissements supplémentaires a été laissé a été lancée en 2018 pour la mandature, s'ajoutant aux 52 centres existants, le projet doit finances pour 2020 prévoit ainsi qu'à 3 millions d'euros en crédits de paiement pour la création de 5 Nouveau Centre par ailleurs une aide à l'investissement de 2 3 millions d'euros permettra de lancer la construction de 5 Nouveau Centre concernant le Centre associatif habilité le développement de ce type de structure apparaît aujourd'hui nécessaire dans un 1er rôle dans un 1er temps afin de fournir à la peau, la justice, une alternative à l'incarcération des mineurs multirécidivistes ou ayant commis des faits d'une grave particulièrement grave en effet développer des alternatives à la prison pour les jeunes délinquants permet de croire et d'espérer que ces jeunes ne connaîtront jamais la prison, certes, les crédits immobiliers concernant les CEF sont clairement intégré dans le PLF 2020, mais l'encadrement des jeunes qui sont accueillis est loin d'être satisfaisant par le manque de postes ou par le nombre de postes vacants ce qui peut nous interroger une autre question doit nous interpeller madame la ministre, celle du nombre de jeunes placés en centre éducatif fermé dont les 2 tiers avaient auparavant été suivie par les services de la protection de l'enfance, une telle proportion conduit à se poser des questions sur l'efficacité de la prise en charge socio-éducative, ces mineurs souvent victimes de carences éducatives et familiales ou livrés à eux-mêmes face à une délinquance de plus en plus précoce, il me semble urgent de mettre autour de la table tous les acteurs de la protection de l'enfance pour la rendent plus efficace, sans jamais oublier, même si ce n'est pas facile que les familles de ces jeunes ne doivent pas être exclus de cette problématique, il conviendra donc de traiter avec beaucoup d'attention cette question au cours des états généraux de l'hébergement, qui vise à réfléchir aux solutions apportées à la situation critique dans les foyers collectifs, les foyers de jeunes travailleurs et les essence d'éducatif renforcés. Merci, la parole est à Madame Josiane Costes pour le groupe RDSE pour 6 minutes. Madame la présidente. Madame la garde des sceaux, mes chers collègues, la mission Justice du projet de loi de finances pour 2020 voit ses crédits cette année encore augmenté de 2 8 pourcent, soit une hausse de 205 millions d'euros supplémentaires par rapport à 2019 au total ce sont 1520 créations de postes qui sont prévues pour cette mission, mission qui se divise en 3 programmes, la protection judiciaire de la jeunesse, sur laquelle je me suis exprimé en tant que rapporteur pour avis de la commission des lois, l'administration pénitentiaire, l'administration pénitentiaire, excusez-moi, et en fait, la justice judiciaire et l'accès au droit, c'est donc sur ces 2 derniers programmes que je concentrerai mon propos : la répartition des crédits se faisant de manière très inégale au profit du programme Administration pénitentiaire, en effet, la grande majorité des postes créés dans ce PLF concerne l'administration pénitentiaire, plus de 1000 créations d'emplois sont prévues, dont 543 correspondent à des postes de surveillants ces recrutements permettront je l'espère, de remédier au problème de la vacance du personnel pénitentiaire et notamment de renforcer les services pénitentiaires d'insertion et de probation mais également d'améliorer les conditions de travail du personnel, un grand effort budgétaire est également fait en matière d'immobilier pénitentiaire, même si nous sommes loin de ce qui était prévu pour les prisons dans la loi de programmation pour 2018, 2022 pour rappel, le gouvernement prévoit de créer 15000 nouvelles places de détention d'ici 2027 et non d'ici 2022 comme annoncé afin d'atteindre l'objectif de 80 pourcent d'encellulement individuel ce projet indispensable pour lutter contre la surpopulation carcérale, bénéficie d'une hausse de 88 millions d'euros de crédits en 2020, satisfaction également qu'un budget de 100 millions d'euros, soit, compte consacré à la crise, construction de 2 prisons expérimentales centrées autour du travail aussi c'est de prison ainsi que les places de structures d'accompagnement vers la sortie les sas dont la construction est également prévue dans le PLF 100 des bons signaux envoyés dans ce sens, s'agissant du programme Justice judiciaire et accès au droit, mon appréciation est plus mitigé mais je tiens aussi à saluer les efforts à cet égard, il faut remarquer que depuis 2017, le renforcement des effectifs des magistrats se poursuit et commence à porter ses fruits en juridiction,

le PLF prévoit ainsi de continuer sur cette lancée, en ouvrant 384 emplois supplémentaires dans la majorité, correspond à des postes de juge pour enfants de greffiers et de juristes, cette hausse des recrutements ne sera certainement pas suffisante, bien sûr, mais il faut l'a souligné, tout en regrettant vivement encore une fois que ces chiffres soient bien inférieurs à ce votée en mars dernier dans la loi de programmation d'autres points ne m'ont pas convaincu à périmètre constant, les crédits pour l'aide juridictionnelle et les frais de justice diminue de près de 14 millions d'euros en 2020, cette baisse se fonde sur des prévisions faites par le gouvernent le gouvernement qui me laisse quelque peu perplexe au regard de nouvelles techniques d'investigation et de plus en de techniques d'investigation qui sont de plus en plus coûteuse, je partage également les doutes de mes collègues s'agissant de la réforme de l'aide juridictionnelle, présenté par les députés, je considère que ce sujet qui touche un aspect essentiel de notre état de droit ne doit pas faire l'objet d'une réforme précipitée au contraire une large concertation, ainsi qu'une étude d'impact sont plus que nécessaire, s'agissant de la protection judiciaire de la jeunesse, je nie bien reviennent prépa je me risque je me réjouis, simplement de la hausse des crédits, mes chers collègues, je conclurai mon propos en rappelant que la politique pénale ne serait du pas à une affaire comptable, vous le savez madame la garde des sceaux le RDSE est attentif à vos réformes, la politique pénale, c'est avant tout une vision et un projet de société pour améliorer la sécurité de nos concitoyens, nous avons des regrets concernant le projet de loi justice nous avons, nous espérons par conséquent que de prochaines initiatives s'agissant notamment de la récidive verront le jour en attendant à raison des réformes en mais avec les quelques réserves que j'ai évoqué les vote des sénateurs du RDSE seront majoritairement. Je vous remercie, merci. Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice, vous avez la parole pour 20 Minutes. Merci beaucoup, madame la présidente, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, merci pour les observations qui ont été formulées 4 chiffres si vous m'autorisez à à commencer mon propos de cette manière, 4 chiffres pour graver au fond l'impact de ce budget 7 milliards 6 une augmentation de 4 pourcent 1520 créations d'emplois supplémentaires, 300 millions d'euros de plus voilà les 4 Schiff essentiels qui caractérisent le budget de la justice pour 2020, ces 4 chiffres répondent à quatre priorité 5, devrais-je dire, d'ailleurs, la réforme de l'organisation judiciaire la nouvelle politique pénale, la transformation du numérique, de la justice, la réforme de la justice pénale des mineurs et l'accès aux droits et aux victimes, donc voilà ce qui caractérise en quelques mots le budget en chiffres et les priorités que nous y attachons je voudrais maintenant à partir de ces éléments-là répondre aux observations que vous avez formulées tout d'abord à monsieur le rapporteur spécial de la commission des finances, Monsieur le Sénateur Lefèvre j'ai bien compris votre propos, vous dites au fond que ce budget n'est pas à la hauteur, car le gouvernement s'affranchit des engagements qu'il a pris devant vous effectivement le budget comporte 153 millions d'euros en moins par rapport à ce que la loi de programmation aurait prévu, j'ai eu l'occasion de m'expliquer devant votre commission commission sur cette moindre progression et les liée à l'immobilier pénitentiaire et je pense qu'elle ne peut pas se rattacher à une forme d'imprévision car je voudrais ici dire que les terrains pour construire, nous les avons la plupart du temps, nous les avons, en revanche, nous n'avons pas toujours l'adhésion soit des autorités locales, soit des populations locales à la construction de ces établissements pénitentiaires c'est un choix que nous avons à faire entre imposer un établissement à des populations ou des territoires qui ne le souhaitent pas en tout cas pas maintenant ou bien tenir compte de ses souhaits dans ces territoires. Donc c'est cela qui explique que nous avons diminué notre programmation pour cette année de la même manière, il y a quelques hypothèses dans lesquelles j'avais eu l'occasion de l'expliquer, les travaux n'avancent pas tout à fait au rythme où nous le souhaitions, les travaux ou en tout cas les opérations précédant les travaux, je parle ici d'appels d'offres qui serait défectueux ou d'études qu'il faudrait compléter parce que nous avons telle ou telle question archéologique a traité qui n'étaient pas initialement prévu, donc tout cela génère des retards, cela ne signifie pas que les crédits ne seront pas là le moment venu mais nous prenons en compte la réalité de l'avancement des opérations immobilières que nous souhaitions promouvoir, nous ne revenons pas sur l'objectif qui a été affichée au moment du vote de la loi de programmation, c'est-à-dire 15000 places supplémentaires en je, vous avez également évoqué, monsieur le rapporteur, la question de la numérisation, souhaitant qu'elle demeure compatible avec un accès physique, je partage complètement votre souhait de ce point de vue-là puisque, bien sûr, nous souhaitons développer les applications numériques dans notre ministère, c'est une exigence, les avocats le demandent et magistral, demandent les greffiers le demande. Pour autant, nous faisons en sorte que dans chaque juridiction, et vous savez qu'elles sont toutes préservé, enfin le mot préserver n'est pas juste d'ailleurs, elles sont toutes conservées dans chaque juridiction, il y aura un service d'accueil unique du justiciable qui permettra d'accueillir physiquement tous les justiciables et de les accompagner dans les démarches qu'ils auront à faire, qu'il s'agisse de l'aide juridictionnelle ou d'autre chose, je rappelle par ailleurs que nous faisons un effort important dans la mise en place des Maisons France service où j'ai souhaité que dans chacune de ces maisons, il y a un conciliateur de justice qui soit présent. Pour là encore pour pouvoir apporter des éléments d'information ou de résolution de litiges pour certains de nos concitoyens, enfin vous avez évoqué la baisse des moyens de l'AJ, si vous le permettez, je répondrai à ce sujet-là, au moment d'un amendement qui interviendra tout à l'heure, je fais donc là ici simplement une réponse formelle, en disant que cette baisse que vous évoquez, elle répond en réalité à ce qui a été constatée dans les dépenses de l'aide juridictionnelle, l'année dernière et que nous avons reporté cette année, vous le savez, également, nous attendons 9 milliards d'euros supplémentaires qui viendront s'ajouter aux chiffres qui ont été présentés, monsieur le rapporteur Détraigne vous avez également évoqué la question budgétaire pour faire valoir que vous ne souhaitiez pas apporter votre soutien, ce budget, vous mettez en avant essentiellement 4 points si j'ai bien compris tout d'abord un effort pour la justice judiciaire que vous n'estimez pas suffisant, j'avoue que c'est un point que j'ai un peu de mal à comprendre dans la mesure où tant le nombre de magistrats qui augmente, que les investissements en matière Immobilier pour la justice judiciaire que le nombre de greffiers, je rappelle, de ce point de vue que l'École nationale des greffes fonctionne à plein régime avec 3 promotions par an, nous ne pouvons pas faire plus en ce moment, nous avons, me semble-t-il, un effort tout à fait important qui est fait en matière de justice judiciaire et donc je ne partage pas votre opinion, vous avez par ailleurs évoqué la question de la baisse de l'aide juridictionnelle, j'ai j'ai répondu un peu à Monsieur le Sénateur Lefèvre je répondrai un peu plus longuement tout à l'heure. Et vous avez enfin évoqué la question de la suppression des postes de juges d'instruction, je reviens sur ce point qui est important, monsieur le sénateur, puisque je voudrais dire ici que ce que nous avons proposé, c'est pas la suppression des postes de juges d'instruction, c'est le regroupement des fonctions de juge d'instruction dans dans des pôles d'instruction pour qu'il y a plus d'efficacité dans l'exercice de cette mission je vous interroge, en effet, pensez-vous vraiment qu'un juge d'instruction qui gèrent moins de 30 dossiers d'instruction par an et qui travaillent en tant que juge d'instruction, peut-être un tiers de temps sur son service, pensez-vous vraiment qu'il y a une plus-Value à ce travail-là, non pas qu'il fasse un travail qui soit qui ne soit pas tout à fait remarquables, ce n'est pas la question, c'est la question globale du traitement de l'instruction et donc je vous interroge : n'y a-t-il pas intérêt, dans ce cas-là, a regroupé fonctionnellement, c'est si ces emplois au sein d'un pôle de l'instruction et je rappelle ici que le regroupement des fonctions n'entraîne pas la suppression du poste de juge, j'ai dit et je me suis engagé là dessus, il y aura le nombre de juges affectés à telle ou telle tribunal ne diminuera pas, parce qu'il y aurait un regroupement. Des fonctions de juge d'instruction, voilà ce que je souhaitais vous dire monsieur le sénateur Détraigne madame la sénatrice Coste alors je ne sais pas laquelle des trois, sénatrice je dois parler je je parle là, ici, à la première, en tout cas, c'est à dire Je parle à monsieur Marc que je salue, je vous remercie d'avoir souligné le chemin parcouru, vous avez toutefois relevé l'incapacité à respecter la trajectoire budgétaire et à ceux-là, je crois avoir répondu, déjà on aurait pourtant aux sénateurs Lefebvre et Détraigne vous avez par ailleurs madame la sénatrice évoquer les questions liées à la protection judiciaire de la jeunesse, je sais que c'est un sujet auquel vous êtes très attaché, qui vous intéresse beaucoup, vous avez évoqué la. Réforme de l'ordonnance de 45 que j'aurai l'occasion de présenter devant vous, puisque vous le savez, je me suis engagé à ce que nous ayons un débat sur ce sujet là, devant le parlement, donc j'espère que nous pourrons l'inscrire, on on dise on a le 1er semestre 2020 ce serait important et vous avez ensuite évoqué plusieurs questions, notamment la question des centres éducatifs fermés, je voudrais simplement dire ici que pour 2020 les centres éducatifs fermés représente 6,8 pour 100 de l'ensemble des coûts alors que l'hébergement collectif est à 25 pourcent les centres éducatifs renforcés 1 pourcent le placement familial et le placement diversifié donc on voit bien que les centres éducatifs fermés, contrairement à ce qui est parfois dit ne représente qu'une partie et pas la plus importante de l'ensemble des autres solutions que nous offrons pour la prise en charge de ces jeunes, je rappelle également que dans les mesures nouvelles, je m'adresse. En disant cela également madame la sénatrice à ceci, qui a relevé ces mêmes problématiques, je rappelle que dans les mesures nouvelles, les centres éducatifs fermés ne représente que 2 47 millions d'euros sur les 11,4 millions d'euros de mesures nouvelles que nous offrons que nous offrons dans le budget 2000. 20. Voilà madame la sénatrice, ce que je souhaitais vous dire, j'ai bien entendu évidemment la question que vous avez évoquées du traitement pénal des mineurs non accompagnés qui est un véritable sujet et mais qui ne peut pas être traité à lui seul qui doit être englobés dans la prise en charge globale des mineurs non accompagnés, puisque ce n'est qu'un des aspects de ce problème de cette question extrêmement singulière. Monsieur le sénateur pu vous avez évoqué la question également des juridictions judiciaires, je cherche sénateur qui a pu, pardonnez-moi, vous avez également évoqué la question des juridictions judiciaires, vous dites que c'est le budget qui augmente le moins je crois avoir répondu en disant répondu en disant que c'est un budget qui, à la fois nous permet de recruter les personnels dont nous avons besoin, qui nous permet de faire de la programmation n'immobilier judiciaire et vous avez également évoqué les crédits qui ont augmenté, il faut le rappeler de 9 pourcent l'année dernière et c'est la raison pour laquelle cette année, nous stabilisons ces mêmes crédits pour prendre en compte l'augmentation qui avait eu lieu l'année dernière et nous les stabilisant à une hauteur à peu près comparables à celles de l'année dernière, vous avez également évoqué la question du recrutement des personnels, nous recrutons les personnels tels que nous nous y étions engagés, donc à la fois des magistrats, des personnels de surveillance pénitentiaire des conseillers d'insertion et de probation de probation 400 cette année, donc je pense que nous aurons l'occasion nous aurons la possibilité ainsi de faire face aux besoins qui sont les nôtres, monsieur le sénateur Sueur vous avez ne posez la question de la comparaison entre le budget de la justice française et et les comparaisons européennes qui sont faites et remarquablement effectués par la C. Paige et mais d'ailleurs aussi par l'Union européenne dont conseil européen et Union européenne. Il n'y a jamais assez d'argent pour la justice, monsieur le sénateur, je vous rejoins aisément sur ce point-là. En revanche, je trouve que les comparaisons doivent toujours être faite avec beaucoup de précision et beaucoup de regards distanciés par exemple je je ne citerai que cela dans les juges en France, nous avons à prendre en compte les juges prud'homaux les juges consulaires, ces juges qui existent dans notre pays ne sont pas comptabilisés dans les études européennes, or ils existent, ils tranchent des litiges, donc ce sont des points qu'il faut réellement prendre en compte, je crois que lorsque l'on veut vraiment comparer et je ne dis pas cela en forme de dédouanement, je dis simplement, sachons de quoi nous parlons, sachons de quoi nous parlons, vous évoquez également des baisses de crédits, monsieur le sénateur, mais lorsque vous évoquez des baisses de crédits ce ne sont pas des crédits, j'ai cru comprendre en vous entendant, mais plutôt des autorisations d'engagement que vous avez évoquée et c'est normal puisque ces autorisations d'engagement ont été ouvertes en 2018, 2019 pour pouvoir lancer toutes les opérations immobilières ou les grands projets informatiques à partir de là, nous sommes en crédits de paiement et donc on ne peut pas comparer, vous le savez fort bien autorisations d'engagement et crédits de paiement, vous avez ensuite évoqué la question des personnes détenues, vous dites au fond, elles sont en augmentation, bon et les mesures alternatives ne sont pas suffisantes, c'est vrai, nous sommes, nous sommes dans une situation difficile en termes de surpopulation carcérale, j'ai quelques espoirs d'amélioration, les tout les tout derniers chiffres montrent une légère baisse des personnes en détention, cette baisse est due, je le crois, aux premières mesures liées à la loi de réforme pour la justice qui, vous le savez, a mis en place dès le 1er juin dernier la libération sous contrainte aux 2 tiers de la peine pour les peines de moins de 5 ans ces premières mesures ont été appliquées et ont connu une augmentation importante, je crois que c'est 90 pourcent d'augmentation de ces premières mesures qui se traduisent d'ores et déjà, mais ce n'est qu'une conséquence sur la question de la surpopulation carcérale, je j'allais dire, je touche du bois, ce n'est pas le mot je ne crie pas victoire, nous sommes dans une politique extrêmement volontariste, une politique de traitement des peines et de traitement des parcours de détention et je pense que tout cela devrait conduire à des améliorations dans quelque temps et sachez par ailleurs que nous sommes extrêmement volontariste pour multiplier les peines autonomes, autre que l'emprisonnement, je pense aux travaux d'intérêt général et je pourrais également parler du bracelet. Enfin, vous avez évoqué la spécialisation des tribunaux, monsieur le sénateur, vous me dites, mais cette spécialisation des des contentieux entre tribunaux lorsqu'il y a plusieurs tribunaux judiciaires dans sa même département, vous me dites ça peut conduire à dépouiller, hein, l'un de ses tribunaux. Mais non, mais non dans la loi, nous avons grandement insisté sur le fait que la spécialisation, c'est une façon de mieux rendre la justice, mais qu'elle devait être équilibrée entre chacun des tribunaux d'un même département, il ne peut pas y avoir d'un tribunal dépouillé par un autre, mais un équilibre qui conduit à une spécialisation des magistrats sur quelques contentieux technique c'est une meilleure justice, ce n'est pas le dépouillage non le dépouillement d'un territoire, pardonnez-moi. Alors sur la question précise que vous que vous m'avez posé, je rappelle que dans la loi, dans la loi telle qu'elle est écrite, nous travaillons sur des propositions de chef des cours d'appel, pas des chefs de juridiction de chefs de cour d'appel et que ces propositions, doit faire l'objet d'un avis des conseils de juridiction, c'est ainsi que la loi est écrite et c'est ainsi que je le respecterai, monsieur le sénateur Soilihi, je vous remercie pour vos propos, j'ai bien entendu pardonnez-moi juste parce que je vois le temps qui s'écoule, j'ai retenu un point précis qui était le numérique Outre-mer je suis extrêmement attentive et c'est un point auquel je veillerai vraiment madame la sénatrice à-ci vous m'avez dit que, au fond, toutes les réformes que nous conduisons ne ferait que allonger les délais de traitement et les délais de traitement des contentieux mais madame la sénatrice, je voudrais simplement vous dire ici que il a déjà été constaté que le délai de moyens de traitement des procédures pénales en matière criminelle, par exemple, est passé de 14 ou de 40 mois en 2017 à 39 en 2019 que le délai moyen de traitement des procédures civiles poursuit sa décrue en 2019, et je pourrais continuer, mais ce n'est pas la peine, car vous allez pouvoir vous reporter à ce document qui n'est autre que celui rédigé par votre commission des finances, et par monsieur Antoine Lefèvre, donc je pense que vous aurez la toutes les réponses nécessaires, madame la sénatrice, notre objectif est évidemment de diminuer les délais de traitement, même si je le reconnais, nous ne sommes qu'au début de cette démarche sur la question de l'éloignement des du des justiciables vraiment non, vraiment non partout les tribunaux restent ils sont même confortés dans l'exercice de leurs compétences et de leur contentieux, je vois que vous dites non, madame la sénatrice, mais j'ai, je ne suis pas en accord avec votre négation, regardez les tribunaux de proximité, madame la sénatrice les tribunaux proximité qui sont tous maintenus et qui pourront voir les contentieux qui sont traités accrue par de nouveaux champs de compétence qui correspondent à la justice du quotidien nous rapprochons le justiciable de ces juges dans la plupart des sites. enfin sur les moyens dédiés à l'enfermement, je vous ai répondu tout à l'heure, les crédits Seif ne sont pas à la hauteur que vous évoquiez, madame la sénatrice vermeil et j'ai entendu vos doutes sur le PNAT brush nous ne partageons pas la même opinion je pense que les résultats du CNAT me permettront vous permettront de constater d'ici quelque temps que le traitement de la lutte antiterroriste et mieux prise en charge du travail de l'intérêt général qui est est du l'insertion professionnelle, d'ores et déjà, on peut constater un véritable engouement pour les travaux d'intérêt général qui en moins d'un an, ont connu une augmentation de plus de 10 pourcent d'offres des postes et davantage de prononcer également je n'irai pas au-delà, simplement je répondrai à j'ai beaucoup apprécié, madame la sénatrice que vous avez dit sur l'humilité et la ténacité, c'est exactement l'esprit dans lequel nous sommes et donc voilà ce que je souhaitais vous dire madame la sénatrice Eustache-Brinio vous avez

rénové, la formation des éducateurs suite à leur passage en catégorie A, qui exige donc un bac plus 3 avec un processus d'alternance intégrative avec des cycles de formation théorique à l'École nationale de la PJJ qui alternent avec des stages pratiques pendant 18 mois plus 4 mois de stages d'accompagnement à la prise de poste, je pense que la formation une formation adaptée, est aussi un moyen d'attractivité dans ses fonctions. Simplement d'un mot pour vous dire que la gouvernance La gouvernance autour de la prise en charge des jeunes par l'ASE sous l'impulsion de mon collègue Adrien taquet sera renouvelé en mettant autour de la table et les juges des enfants et les départements et la PJJ et là, The pour qu'on ait vraiment qu'on essaie d'avoir une prise en charge plus coordonnées, vous avez parfaitement raison de souligner madame la sénatrice Coste je m'adresse à nouveau à vous pour vous dire que les la question des personnels pénitentiaires et notamment des vacances des personnels pénitentiaires, juste un un mot là-dessus, nous travaillons beaucoup sur ses vacances, des personnels pénitentiaires et des surveillants pénitentiaires avec des primes pour donner davantage d'attractivité à ses fonctions et avec une redéfinition des postes plus large pour avoir une carrière plus attractive, merci en tout cas, mesdames et messieurs les sénateurs, de vos propos. Merci madame la ministre, nous avons procédé à l'examen des amendements portant sur les crédits de la mission Justice figurant à l'état B article 38 crédits de la mission, nous avons l'amendement 893 présenté par le gouvernement. madame la ministre, place Vendôme, bien sûr, le site historique et sur un nouveau site, porte d'Aubervilliers, dans le 19ème, le site du millénaire c'est ce site-là, qui regroupe le plus d'agents, il abrite le site du millénaire, les services du secrétariat général de la direction des services judiciaires, de la direction de l'administration pénitentiaire et de la direction de la PJJ, ainsi que l'inspection générale de la justice, et compte tenu des créations d'emplois récentes et à venir, notamment en matière du développement numérique du développement de plan de transformation numérique et du renseignement pénitentiaire, nous avons besoin de trouver de la place et donc le départ de l'ARS d'Île-de-France d'un bâtiment tout à fait voisin, celui que nous occupons actuellement nous semble être une opportunité et donc nous avons un projet d'installation des services de la chancellerie dans les espaces qui sont actuellement loués par l'ARS, mais nous manquons d'autorisations d'engagement pour signer le bail, la loi de finances initiale pour 2019 a prévu un montant de 41 millions d'euros en autorisations d'engagement au bénéfice du programme 310 cette budgétisation correspondait à à l'hypothèse à l'hypothèse initiale d'un engagement d'une durée de 6 ans, or le recueil des règles de la comptabilité budgétaire de l'État, modifié à l'été 2019 prescrite désormais d'engager la dépense à hauteur de la durée totale du bail et donc nous voyons-nous, comme nous voulons un bail de 9 ans dont 7 ans ferme le montant des autorisations d'engagement s'élève à 54,3 millions d'euros, c'est la raison pour laquelle on a besoin d'un financement complémentaire de 12,4 millions d'euros que je vous serais reconnaissant de bien vouloir accepter. Merci, quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Alors sur le fond, il y a pas de difficulté madame la garde des Sceaux, par contre, sur la forme comme tenu de la décision de rejet des crédits, ce sera un avis défavorable. Merci, y a-t-il des demandes d'explications de vote, il y en a pas, je vais donc mettre aux voix l'amendement 893 avec un avis défavorable de la commission qui est pour. Qui est contre, il n'est pas adopté un amendement 698 Madame la ministre. la loi de 2014 sur la formation professionnelle prévoit que vous le savez, que la région est désormais l'acteur clé de la formation professionnelle et l'acteur unique, l'article 61 21 tiré 2 du code du travail, dispose que la région finance et organise la formation professionnelle des personnes sous main de justice, il prévoit également la conclusion d'une convention entre l'État et les régions qui précise les conditions de fonctionnement du service public régional de la formation professionnelle au sein des établissements pénitentiaires, un transfert du programme 100 cette administration pénitentiaire est intervenu en loi de finances initiale 2017 pour un montant de 490000 euros pour compenser financièrement la reprise de la compétence, par les régions, ce transfert, porter sur la masse salariale afférentes aux missions transférées le ministère de la justice, conservant les effectifs assurant au niveau des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, le pilotage des actions d'accueil d'orientation et d'évaluation de la population pénale le présent amendement correspond à un ajustement technique visant à prendre en compte le besoin du département de Mayotte. Merci, quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Alors, même si c'était bien tenté, madame la garde des Sceaux et effectivement, vu les sommes en jeu, ce n'est pas pour les les 10000 euros, que cela concerne, on était toujours d'accord, on peut être d'accord sur le fond, mais compte tenu du rejet des crédits, ce sera encore un avis défavorable. Très bien, il n'y a pas de demande d'explication de vote je mets aux voix l'amendement 698 avec un avis défavorable de la commission qui est pour. Qui est contre.

Merci, présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, je me félicite du lancement de la construction du centre de détention de dans les travaux vont pouvoir commencer en 2020, l'ouverture de ce centre va permettre de désengorger le centre pénitentiaire de Nouméa, mais les locaux du commerce sont particulièrement vétustes et ce qui renforce l'insécurité dans ce centre, je propose donc de prévoir dans ce budget, une enveloppe de 40 40 millions d'euros sur 4 ans pour rénover le connaissent et ainsi améliorer la sécurité du personnel pénitentiaire et les conditions de détention des prisonniers. Merci, quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur, avis défavorable, défavorable, Madame la Ministre. Pardon. Oui, mais ma vie, je m'explique simplement Monsieur le Sénateur, en 2 mots, nous en sommes actuellement au centre de Nouméa sur la question des études, la direction de l'administration pénitentiaire est en train d'étudier les différentes études et les différents scénarios de réhabilitation qui ont été proposées, qui suppose, bon enfin ces différents scénarios, donc nous n'avons pas besoin sur le budget 2020 de mettre en place des financements, puisque ces études seront prises en charge sont les crédits dont nous disposons déjà en revanche, comme vous le savez, vous l'avez rappelé le centre de connaît, lui dont les travaux commencent, si je ne me trompe pas ce mois-ci pourra ouvrir comme prévu en 2021 mais donc nous n'avons pas besoin en 2020, d'un financement sur le Centre pénitentiaire de Nouméa. Merci oui, explications de vote, mais c'est sur. Oui merci madame la présidente, la vie de la de la commission est défavorable parce que la commission est défavorable sur cet amendement ou par rapport à la logique générale de rejet des crédits de cette mission, s'agissant d'une question très importante soulevée par par notre collègue est ce que je pourrais avoir plus de précisions de la part de la Commission.

le vote est très serré, donc je vais vous demander de relever la main à nouveau.

L'amendement est adopté. Nous passons à l'amendement 896 rectifié Madame Coste. Merci madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, le financement de l'aide, je dirais juridictionnel et l'une des problématiques rue qui récurrente intéressant, le ministère de la justice qui pose la question de l'accessibilité financière à l'État de droit, quel intérêt en effet de consacrer des droits pour protéger les individus les plus vulnérables de notre société, si dans le même temps, le coût d'entrée dans le système judiciaire les empêche de les faire respecter en moderne à la nécessité d'offrir aux personnes démunies, une aide juridictionnelle, a été reconnu depuis 1851 si l'existence de cette aide n'est pas sérieusement remise en question son périmètre d'application peu l'objet de discussions constantes, comme en témoignent les récentes modifications à la loi du 10 juillet 1991 introduite à la suite du rapport des députés Gosselin et Moutchou celui-ci fait d'ailleurs écho aussi au rapport de 2014 de Sophie Joissains Jacques Mézard, se pose en effet dans ce domaine, comme ailleurs, la question de la soutenabilité du système avec les croissants, l'accroissement des inégalités en France, il est dommage que cette question soit traitée législatives de manière incidente, alors que le sujet mériterait à lui seul un texte spécifique, en l'absence d'un consensus entre les 2 chambres, il nous paraît nécessaire de garantir son financement jusqu'à ce qu'une réforme pérenne satisfaisantes, voit le jour à cette fin, le présent amendement vise à accroître les crédits alloués au programme accès au droit et à la justice afin de renforcer la capacité de financement de l'aide juridictionnelle à partir des besoins de financement identifié par nos rapporteurs je vous remercie. l'avis de la commission, ça serait un avis favorable aussi sur le fond, compte tenu également de ce que le rapport triste Josiane Costes tout à l'heure, a indiqué sur la PJJ, mais là aussi, on sera obligé sur la forme de rejeter les deux rejeter les crédits et donc de donner un avis défavorable. Merci, Madame la Ministre. Merci madame la présidente, c'est également un avis défavorable Madame Cosse, que j'aimais l'amendement que vous proposez, vous proposez par cet amendement d'accroître de 9 millions d'euros, le budget alloué à l'aide juridictionnelle, les 484 millions d'euros de crédits inscrits dans le projet de loi de finances couvre en fait notre prévision de dépenses pour 2020 si les crédits n'augmente que de 61 millions d'euros en 2020, c'est en fait pour des raisons techniques, d'abord cela résulte d'un apurement de enfin, il y a un apurement pardon de produits de contribution pour l'aide juridique, qui restait sur un compte d'attente et qui, je le disais tout à l'heure sera réalisée d'ici la fin de l'année et qui apportera 9 millions d'euros de ressources supplémentaires pour le financement de de l'aide juridique, il y a ensuite une révision à la baisse de l'évolution tendancielle de la dépense d'une vingtaine de millions d'euros, qui a été réalisé au vu de la dépense effectivement constaté en 2018 qu'qui n'étaient que de 464 millions d'euros, nous prévoyons en outre par sécurité de reporter les crédits du programme 101 accès au droit et la justice qui ne seront pas consommés en 2019 sur l'aide juridictionnelle, ça devrait représenter à peu près 13 millions d'euros pour autant la dotation inclut une enveloppe de 4 millions et demi d'euros pour financer l'extension de la représentation obligatoire qui est prévu dans le d'un texte qui va sortir dans quelques jours, ainsi que 5 millions d'euros pour développer la contractualisation avec les barreaux et financé notamment l'expérimentation dessus 2 structures dédiées à la défense des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, j'émets donc un avis défavorable. Merci donc nous avons 2 avis défavorables qui est pour. Qui est contre, n'est pas adopté l'amendement 898 président requis

Commission européenne pour l'efficacité de la justice, il a découvert ça tout à l'heure, alors les moyens humains, sur la manière, la matière première, la justice, du début à la fin de la chaîne judiciaire je ai pas ce magistrat, évidemment, mais également au greffier, agent administratif chargé de les assister dans leurs missions régaliennes à nous et nous nous inquiétons doit appliquer au monde judiciaire comment d'autres domaines avant lui un fétichisme électronique qui consisterait à penser que les peuvent trouver des solutions pérennes et acceptable, il y a des algorithmes informatiques,

paradoxalement le déficit d'investissement a conduit notre juridiction a développé une productivité hors norme pour maintenir des, des, des jugements qui soit qu'il table après les sanctions des juges européens et afin de maintenir un accueil digne des justiciables locaux parfois très détériorée, de la justice, nous, nous, nous ne sommes pas de votre volonté devrait signer significativement en rentrant pas le Français à la matière et l'option de la loi de programmation cette année année la première manifestation toutefois au regard des engagements fixés par cette loi, nous considérons une autre motivation des crédits est possible afin d'accompagner ce rattrapage est d'abord et d'améliorer oui en substantielle le service public de la justice dans pays les amendements donc à prolonger l'esprit de la loi de programmation et à proposer des transferts de crédits notamment des postes informatiques vers les juridictions afin d'y renforcer la présence humaine. Merci, monsieur le rapporteur, c'est à vous pour l'avis de la commission. Avis défavorable pour les raisons indiquées précédemment. Merci madame la ministre. Merci madame la présidente, c'est aussi un avis défavorable, mais je voudrais dire à monsieur le sénateur, qui est que je suis évidemment extrêmement sensible à l'argumentation qu'il a développé, je voudrais vous dire monsieur le sénateur, qu'on a fait en 2020, un effort important pour les services judiciaires puisque, en réalité, nous créons 384 emplois en 2020, 384 emplois qui se décompose en 100 emplois de magistrats et 284 emplois de personnels de greffe et d'assistés de juristes assistants et de fonctionnaires, c'est sans emploi de plus que ce qui était prévu dans la loi de programmation donc sur ce point-là, nous avons fait un effort supplémentaire par rapport à ce qui était prévu dans la programmation, c'est un effort supplémentaire qui est ciblé, j'ai eu l'occasion de le dire, puisque sur l'ensemble de ces emplois, nous allons essentiellement accompagnée de politique prioritaire la réforme de l'ordonnance de 1945 sur la justice pénale des mineurs, avec 70 emplois de magistrats et puis sans greffier et puis également des personnels PJ, mais mais non, je ne parle pas ici et puis le 2ème, le 2ème Champ sur lequel j'interviendrai positivement, c'est les au sein de la des juridiction interrégionale spécialisée pour lutter contre la délinquance et notamment la délinquance financière, qui me semble devoir être également une de nos priorités 30 magistrats et des personnels supplémentaires, on a des personnels plus que ce qui était prévu dans la loi de programmation et nous les affectons sur 2 politiques prioritaire, pour autant, je ne dis pas que tout va bien, d'une part nous devons retravailler sur notre grille d'affectation des magistrats sur notre ce qu'on appelle notre clé de répartition des magistrats, la direction des services judiciaires s'y attache, et c'est un projet qui arrivera à terme dans un ou 2 ans, et d'autre part, nous devons également prendre en compte des emplois pour la réforme du. Contentieux social puisque, vous le savez, nous avons mis en place l'année dernière, la réforme du contentieux social et de ce point de vue là il y a 132 emplois qui seront transférés du ministère de la Santé et des solidarités, pour nous aider à prendre en charge contentieux sociales donc voilà un effort important, bien sûr, qui demande à être poursuivi, mais c'est un effort particulièrement important que nous faisons pour cette raison, j'émets un avis défavorable à votre amendement monsieur. Merci et donc mettre aux voix l'amendement 890 Monsieur Ruquier.

Merci madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le 6 novembre dernier nous avons adopté la proposition de loi visant à agir contre la violence au sein de la famille, ce texte prévoit de généraliser l'utilisation du bracelet antirapprochement afin de mieux protéger les victimes de violences conjugales, c'est un dispositif attendu et qui a fait ses preuves dans plusieurs pays européens, je crois qu'il est temps de passer de la parole aux actes en inscrivant dans ce budget, les 5,5 millions d'euros nécessaires à la mise en place du bracelet antirapprochement je rappelle aussi que ce bracelet devra bénéficier à tout le territoire, y compris à la Nouvelle-Calédonie, qui est particulièrement touchée par les violences conjugales, je rappelle que je viens de déposer un amendement parce que, effectivement, il y a une nécessité de rénover le camp hein ça parce que il y a, il y a un surplus de prisonniers et on a des difficultés, non moi je, je demande à ce qu'il y a un effort de fait pour éviter qu'on ait des prisonniers en plus merci. Merci, quel est l'avis de la commission. Oui, Madame la Ministre. Monsieur le sénateur, j'aime également un avis défavorable à votre amendement, bien que j'en partage l'objectif, vous avez raison il faut sur ce Champ-là absolument passer de la parole aux actes, mais j'estime précisément que le dispositif financier que nous avons construit va nous permettent de passer de la parole aux actes sur les bracelet antirapprochement je me suis engagé à ce que nous en déployant 1000 en 2020 pour ce faire, c'est l'administration pénitentiaire qui prendra en charge ce déploiement, l'administration pénitentiaire qui assure d'ores et déjà, le suivi du placement sous surveillance électronique mobile pour les personnes qui sont placées sous main de justice. Plusieurs marchés sont nécessaires pour mettre en oeuvre le bracelet antirapprochement plusieurs marchés un marché négocié sans mise en concurrence avec le prestataire actuel du bracelet électronique pour adapter le système saphir qui est le système actuellement utilisés, d'une part et d'autre part, un marché pour la fourniture des bracelets eux-mêmes, qui est un marché de téléassistance, qui feront l'objet d'appels d'offres et donc on est en train de définir le cahier des charges, je sais presque terminé et les modalités de fonctionnement du dispositif, le coût de cette mesure en 2020, il est estimé comme vous l'avez rappelé entre 5 et 6 millions d'euros, je ne peux pas dire précisément puisque ça va dépendre des appels d'offres et des marchés qui ne sont pas passés ce coup, je vous le dis, il est pris en charge par le programme 107 de l'administration pénitentiaire, grâce à un report de crédits de 6 millions d'euros de l'exercice 2019 sur 2020 et ce report de crédits il est inscrit dans la loi de finances rectificative qui va vous être présenté d'ici quelques jours et vous en trouverez la la traduction, il n'est donc pas utile de. Revoir à ce stade un abondement du programme 107 comme vous le proposez, c'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable. Merci madame Darcos vous avez la parole. remercie beaucoup notre collègue parce que je pense qu'à un moment donné, il faut que, symboliquement, ça soit fléchée, vous dites qu'on va la voir dans le rectificatif je j'imagine que cet amendement peut-être ne n'ira pas jusqu'au bout, mais évidemment de l'approche du projet loi de finances, mais on a eu cette discussion, vous vous souvenez, déjà sur le fait que peu de juge des affaires familiales n'osez entraver la liberté d'un dans d'un mari battu et donc c'était pas forcément impliqué qu'il fallait plutôt partir, partir sur un juge des libertés et de la détention mais honnêtement le budget même du bracelet est en effet extrêmement coûteux, comme vous l'avez dit je vous fais confiance mais je vais voter l'amendement de mon collègue parce que, honnêtement, que rien n'était fléchée en tant que telle dans cette loi de finances, alors que ça fait moins de 3 semaines qu'on a voté cette proposition de loi sur ces, sur ces bons, ça me paraît inconcevable vis-à-vis des familles vis-à-vis des des victimes si vous peut-être que symbolique, mais pour moi c'est très important. Merci, il n'y a pas d'autres demandes de parole bien, je vais donc mettre aux voix l'amendement 297 avec 2 avis défavorables qui est pour. 5 6 7 6. Qui est contre. Il est adopté. Nous allons procéder au vote des crédits de la mission Justice figurant l'état B je n'ai été saisi d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite je mais on voit les crédits de la mission, j'ai j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe LR sur les crédits de la mission Justice inscrite à l'état B. Il doit être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement, le scrutin est ouvert.

Très bien, le plus personne ne demande à voter, le scrutin est clos. J'invite les secrétaires et constater les résultats du scrutin. Voici

Voici le résultat du scrutin numéro 56 compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordé par les sénateurs aux groupes politiques et notifié à la présidence Nombre de votants : 341 Nombre de suffrages exprimés 333 pour l'adoption 42 contre 291 le SIDA n'a pas adopté.

parce que vous avez un nombre de vous pas supérieur au nombre de voix contre. Voilà donc article 76, terre des siestes, nous avons 2 amendements identiques les amendements de suppression d'amendement 22 présenté par Monsieur Lefebvre. Oui, madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, cet amendement vise à supprimer la réforme de l'aide juridictionnelle, dont on a déjà beaucoup parlé, proposé par le présent article qui traduit une partie des préconisations du rapport de la mission d'information sur l'aide juridictionnelle menées par nos collègues députés Naïma Moutchou et Philippe Gosselin alors qu'actuellement le demandeur de l'aide juridictionnelle doit justifier que ces ressources mensuelles sont inférieures à 1000 euros pour l'aide juridictionnelle totale et à 1500 euros pour l'aide juridictionnelle partielle et que les bureaux d'aide juridictionnelle doivent tenir compte des ressources de toute nature dont dispose le demandeur, il est proposé de tenir le revenu fiscal de référence comme critère d'éligibilité, afin de garantir une application équivalent de ce critère partout, les bureaux d'aide juridictionnelle, or l'article renvoie la définition des plafonds annuels d'éligibilité à l'aide juridictionnelle, un décret en Conseil d'État, alors même que les plafonds actuels sont actuellement prévus par la loi, ce qui ne permet pas au Parlement d'évaluer les impacts de la mesure proposée, notamment s'agissant de la population éligible à l'aide juridictionnelle, de même les modalités d'estimation du Patrimoine et des ressources imposables à prendre en compte lorsque le revenu fiscal de référence n'est pas applicable sont renvoyées à un décret de plus alors qu'un bureau d'aide juridictionnelle est actuellement établi au siège de chaque tribunal de grande instance l'article prévoit que le bureau d'aide juridictionnelle sera désormais établie au siège des juridictions, dont la liste est le ressort en cette matière seraient définies par décret prévoit donc la suppression de certains bureaux d'aide juridictionnelle et renvoyant leur localisation et la voie réglementaire, enfin, aucune étude d'impact n'accompagne ces propositions car cet article résulte d'un amendement portant article additionnel voté par l'Assemblée nationale, ainsi pour toutes ces raisons, il y a lieu de supprimer cet article. Merci, nous passons à l'amendement 514 Monsieur Détraigne. C'est le même amendement il est défendu. Si Madame la Ministre. Merci madame la présidente, votre amendement, messieurs les sénateurs, vise à supprimer les éléments de réforme de l'aide juridictionnelle, tels qu'ils ont été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, que je suis peut-être un peu gênée par l'un des arguments que vous avez avancés, à savoir celui de l'absence d'étude d'impact, cet amendement, vous l'avez souligné vous-même, il est d'origine parlementaire, c'est un amendement qui a fait suite au rapport qui a été élaboré par Madame Moutchou et par monsieur Philippe Gosselin, député, il a donc été adopté par ailleurs de manière complètement transpartisane à l'Assemblée nationale, les amendements parlementaires, vous le savez, ne nécessite pas d'étude d'impact et à suivre votre raisonnement en invoquant cette irrégularité au fond vous semble riez considérer que les parlementaires ne peuvent pas porter d'études et de réformes ambitieuses à la suite d'un véritable rapport qui au fond sert en lui-même d'étude d'impact, je suis donc un peu étonné de cette démonstration au demeurant l'incidence financière de cet amendement sera relativement faible, l'objectif est de fixer l'aide juridictionnelle en référence, vous l'avez rappelé au revenu fiscal de référence, il ne devrait pas modifier sensiblement le périmètre actuel des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, il comporte par ailleurs des mesures d'économie, je ne partage pas non plus Monsieur le Sénateur, Lefèvre, votre 2ème enfin, l'un des ours, argument qui a été avancé, selon lequel les plafonds devraient être fixé dans la loi les plafonds d'admissions à de très nombreuses aides sociales sont d'ores et déjà fixé par le pouvoir réglementaire, c'est par exemple le cas des aides au logement du revenu de solidarité active et je pourrais en citer d'autres encore le pouvoir réglementaire peut donc fixer des montants de plafond de ressources ouvrant droit à certaines aides comme les allocations logement, dès lors que la loi en fixe le cap et l'article qui est adopté par l'Assemblée nationale fixe clairement l'objectif : les limites et les correctifs à prendre en compte pour prendre pour octroyer l'aide juridictionnelle. Enfin, s'agissant du dernier point que vous avez évoquées, à savoir la nécessité de maintenir un bureau d'aide juridictionnelle au sein de chaque tribunal judiciaire dans la loi, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la réalité, un très grand nombre de bureau d'aide juridictionnelle sont gérés par une une ou 2 personnes et donc garantir la continuité du service, la qualité du traitement des demandes, la durée de l'instruction, c'est extrêmement difficile dans de nombreuses juridictions donc dans ce contexte, il n'apparaît pas anormal que j'législateur octroie aux pouvoirs réglementaires, la capacité de mieux organiser les circuits d'instruction de l'aide juridictionnelle afin d'éviter, donc des situations dans lesquelles l'absence d'un agent peut mettre en péril le bon fonctionnement d'une juridiction, mais contrairement à ce que vous semblez redouter cette disposition comme d'ailleurs la précédente sur la question des critères de ressources, ouvrent la perspective d'un octroi beaucoup plus rapide et beaucoup plus sécurisé de l'aide juridictionnelle, ce qui permettra de répondre bien mieux qu'aujourd'hui, à l'urgence en matière pénale, ça ne signifie pas qu'il n'y aura plus de contacts de proximité pour le justiciable, j'ai eu l'occasion de vous répondent dans mon propos introductif, le service d'accueil unique du justiciable dans chaque juridiction et là pour cela, il pourra évidemment accueillir les dossiers et répondre aux questions qui seront formulées mais avec un système informatique nationale performants comme celui que nous voulons créer qui pourra donc contrôler automatiquement le revenu fiscal de référence, l'instruction de la demande d'aide juridictionnelle pourrait être organisé différents différemment de la manière dont elle est aujourd'hui, nous travaillons d'ailleurs actuellement avec six juridiction. Pilote pour définir la meilleure organisation donc pour ces raisons, je regrette que vous ne n'approuvait pas ces dispositions qui, je ne crois vont pouvoir prendre le dispositif d'aide juridictionnelle, plus efficace et plus performant et j'émets donc un avis défavorable sur merci Monsieur Bonhomme, vous avez la parole. Merci, mais dans la présidente oui, moi aussi, dans le même sens, c'est mon amendement suivant : effectivement, je pense que l'étude d'impact aurait été favorable alors vous dites, madame la ministre, que ça a été transpartisan mais je ne vois pas en quoi ça viendrait invalider le fait qu'une une évaluation, peut-être sous la forme d'étude d'impact aurait été nécessaire pour une telle décision et je pense que l'amendement de suppression qui est proposé ici à l'Avantage de revenir à de

au demeurant le le maintien des bâches dans l'état actuel au sein des TJ, me paraît vraiment le lieu, le lien pertinent pour tenir compte du lien propres, qu'il y a entre les TGI et le barreau et en encore, c'est particulièrement vrai en matière pénale, puisque le fonctionnement des juridictions et dans ce cas-là particulièrement dépendant des pratiques en matière juridictionnelle puisqu'il faut maintenir ce lien étroit entre notamment le président du tribunal, le procureur, le bâtonnier et son bureau des affaires des

me paraît aussi logique, ce qui aurait permis d'avoir une étude d'impact, je considère à nouveau que l'estimation du coût de cette mesure est important pour décider pleinement de de l'efficacité de cette réforme. monsieur Sueur, vous avez la parole. Merci madame la présidente, madame la Ministre, je partage ce qui vient d'être dit par monsieur Lefebvre, ici au Sénat, nous avons beaucoup réfléchi à la question de l'aide juridictionnelle, je ne sais pas combien de rapports savons fait

que la réforme de l'aide juridictionnelle, qui aurait un sujet c'est un sujet essentiel très important arrive comme ça, en pleine loi de finances, par un amendement de l'Assemblée nationale sans prendre aucunement en compte les réflexions du Sénat qui ont été très approfondie sur ce sujet nous paraissent être sur le plan de la méthode n'être pas satisfaisant de la même manière, vous le savez, nous n'avons pas été ravis d'apprendre que la justice des mineurs seraient réformer par ordonnances, certes, il s'agit d'une ordonnance, je sais, mais nous serons très vigilants et j'espère que Madame la Ministre, vous l'avez dit qu'il y aura un profond débat avant l'adoption des mesures mais pour revenir à cette question de l'aide juridictionnelle, nous, nous avions déposé 3 amendements mais bien entendu, nos 3 amendements, il voit exactement dans le même sens, avec des moyens différents, que les amendements de Monsieur Lefebvre et de Monsieur en effet, nous pensons qu'il y a un vrai problème quant à la prise en compte des ressources prendre le revenu fiscal, ce n'est pas prendre en compte l'ensemble des revenus, deuxièmement, nous sommes attachés à ce qu'il y a un bureau d'aide juridictionnelle dans chaque tribunal de grande instance, même si cela peut susciter des difficultés : attention, attention à éloigner. Le lieu où cela sera décidé de nos concitoyens qui viennent demander de l'aide juridictionnelle, et enfin le fait que le bureau d'aide juridictionnelle pourra refuser des mesures qui paraîtront ne pas pouvoir être acceptée ouvre une porte à l'arbitraire, donc vraiment, nous sommes déçus, nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet de serions vraiment dû être associés à cette réforme, nous pensons que celle-ci a été faite trop rapidement quels risques tente de d'engendrer des conséquences très défavorable, un certain nombre de nos concitoyens, c'est pourquoi c'est dans cet esprit que notre groupe soutiendra les amendements de suppression puisqu'ils sont exactement ils ont exactement le même objet que les trois amendements que nous avons pour notre part déposé. Merci, il n'y a pas d'autres demandes de parole, je vais donc Petro voix l'amendement 22 et l'amendement 514 amendements identiques avec tous 2 un avis défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Ils sont à adopter les 5 amendements suivants tombe et l'article 76, terre des sièges et donc supprimer mes chers collègues, je vais lever la séance prochaine séance ce vendredi 6 décembre à 9 heures 30 pour l'examen de la mission Travail et emploi, oups, du projet de loi de finances pour 2020 la séance est levée.